La séance est reprise. La parole est à M. Bernard Jomier, pour un rappel au règlement.

De plus, nous nous trouvons dans des circonstances particulières et, ainsi que nous l'avons dénoncé, il n'y a pas eu de loi de financement rectificative de la sécurité sociale depuis le début de la crise sanitaire, alors que nous en sommes au quatrième projet de loi de finances rectificative.

qu'à transformer le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) en fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS), il en modifie ainsi le champ comme les dépenses éligibles. s'agit bien d'une concrétisation du Ségur que l'on nous demande de mettre en oeuvre, concernant, notamment, les 6 milliards d'euros d'investissements structurants promis pour la santé, pour l'hôpital, mais aussi pour le secteur médico-social. Or force est de constater que, sur ces éléments financiers qui sont pourtant le nerf de la guerre, l'étude d'impact du PLFSS est relativement imprécise, voire parfois contradictoire. quelques éléments qui ont pu nuire, à mon sens, à la clarté des débats. Le FMIS ne portera pas les 6 milliards d'euros d'investissement, mais 3,9 milliards d'euros. La ventilation de ce grand plan entre les trois grands piliers que sont la santé, le numérique et le médico-social ne reprend néanmoins pas totalement ce qui relève du FMIS. En outre, l'assurance maladie, contributeur du FMIS, continuera d'apporter une dotation annuelle au-delà du Grand plan, mais les fonds que la CNAM apportera, au titre des 6 milliards d'euros, seront, quant à eux, remboursés par l'Union européenne, à travers le plan de relance européen. L'assurance maladie sert donc d'avance à des crédits du plan de relance européen. Nous considérons que cela est original, pour ne pas dire mal venu. On nous promet un fonds transversal visant à lancer des passerelles entre la ville et l'hôpital, entre le sanitaire et le médico-social. Soit, nous signons. Le Grand plan d'investissement contient lui-même, toutefois, trois sous-enveloppes qui distinguent bien entre sanitaire et médico-social. Bref, vous l'aurez compris, si nous soutenons l'effort massif fait en destination des investissements de modernisation de la santé, nous sommes circonspects quant à la feuille de route financière qui nous est présentée. Je tenais à le souligner. J'en viens à l'amendement déposé par notre commission, laquelle a souhaité, sur cet article au dispositif purement juridique de constitution du fonds, s'intéresser davantage à la gouvernance de celui-ci. Nous entendons le souhait du Gouvernement que cette gouvernance soit territorialisée et nous attendons que les contours du futur Conseil national de l'investissement en santé (CNIS) soient précisés. La commission a ainsi souhaité inscrire dans la loi le rôle général du CNIS. Notre préoccupation est bien que la future stratégie d'investissement en santé s'appuie sur les territoires, et, au-delà de la composition du CNIS, nous entendons que la feuille de route nationale appuie des priorités locales et tienne compte des spécificités de certains de nos territoires,

En outre, l'exclusion des cabinets libéraux hors CPTS, équipes de soins primaires et équipes de soins spécialisés, aurait pour conséquence le ralentissement de la modernisation des systèmes d'informatisation en médecine de ville et n'encouragerait pas les médecins à s'investir dans la synthèse du volet médical. Cet amendement vise donc à rétablir cet équilibre. Les

les centres de santé et les maisons de santé. Certains des amendements visant à l'intégration de ces structures sont donc satisfaits sur ce point. La suppression des références vise à élargir le champ des structures d'exercice coordonné. Il s'agit, ici, de prévoir l'éligibilité des cabinets libéraux au FMIS. Je partage cette préoccupation : beaucoup de cabinets libéraux font aujourd'hui des efforts et investissent pour répondre aux besoins en matière de numérique ; notre intention est bien de fluidifier l'usage du numérique à tous les niveaux de la prise en charge du patient. Je suis donc favorable à ce que le fonds leur soit accessible. Je peine, en revanche,

Les autres investissements seront prioritairement dédiés à la transformation, à la rénovation et à l'équipement des établissements médico-sociaux, pour 2,1 milliards d'euros, aux projets hospitaliers prioritaires et investissements ville-hôpital, à hauteur de 2,5 milliards d'euros, ainsi qu'aux enjeux sur le numérique, pour 1,4 milliard d'euros. Il ne s'agit malheureusement pas du premier plan de relance. Je vous rappelle qu'en 2012, qui ont été consacrés à l'hôpital. Pourtant, nous rencontrons toujours des difficultés. La répartition de ces aides à l'investissement sera, pour la plus grande part, pilotée au niveau régional en accord avec les objectifs des projets régionaux de santé et sur la base de critères définis par les Compte tenu des enjeux majeurs que représentent les chantiers visés par ces aides et du caractère particulièrement structurant de ceux-ci pour l'offre de soins, il convient de garantir aux acteurs une visibilité du dispositif. À cette fin,

de la commission ? Cet amendement vise à préciser les modalités d'examen et de sélection des demandes de financement adressées au FMIS. Je soutiens le principe selon lequel il ne doit pas être tenu compte de l'ordre d'arrivée des demandes, ainsi que la nécessité de leur motivation. Je doute, en revanche, de l'opportunité de l'inscription de ces modalités dans la loi. En outre, les rôles du directeur de l'ARS et du comité consultatif d'allocation des ressources tels qu'ils apparaissent dans cet amendement me semblent trop contraignants, alors que les dispositions concernant ledit comité ne sont pas encore stabilisées. Aussi, il me paraît plus pertinent de laisser au champ réglementaire la compétence de précision des modalités de traitement et de sélection des demandes. L'avis est donc défavorable.

M. Martin Lévrier. L'alinéa 10 du présent article vise à permettre aux établissements publics de santé de refuser le paiement des factures de leurs prestataires informatiques lorsque les référentiels d'interopérabilité ne sont pas respectés. L'objectif d'interopérabilité des logiciels en santé est partagé par tous ; celle-ci constitue d'ailleurs une condition au financement des dépenses engagées dans le cadre du volet numérique du FMIS. Il convient ainsi de s'assurer- c'est important ! -du respect des exigences d'interopérabilité des logiciels, lesquelles doivent être intégrées par les professionnels et les structures dans leur stratégie d'achat et comme critères dans les cahiers des charges d'achat de logiciels, avant tout paiement. En permettant aux établissements de s'exonérer du paiement de leurs factures de logiciels, l'alinéa discuté paraît redondant avec les dispositifs déjà prévus et, surtout, contraire aux principes de la commande publique, dans la mesure où il va à l'encontre d'une relation contractuelle existante entre l'établissement public de santé et son prestataire. L'amendement permet d'inscrire le secteur médico-social comme bénéficiaire de ses actions. Aussi proposons-nous d'étendre la faculté accordée aux établissements de santé de refuser le paiement de factures pour non-respect des référentiels d'interopérabilité au champ médico-social, cette garantie ayant la même importance pour les deux secteurs.

un ajout de l'Assemblée nationale ouvrant un droit de refus de paiement des factures dans le cas où les logiciels commandés ne satisferaient pas aux conditions d'interopérabilité. J'avais émis des réserves, dans mon rapport, quant à la conformité de ces dispositions au regard du droit de la commande publique et du respect des obligations contractuelles.

Cette possibilité, dénuée de validité juridique, permettrait de revenir sur une relation contractuelle entre un établissement et son prestataire. C'est en amont de la délibération, de l'élaboration du cahier des charges et de la conclusion du contrat que les établissements doivent exiger l'interopérabilité.

Le Ségur de la santé a prévu la disparition du Copermo au profit d'un Conseil national de l'investissement en santé (CNIS) qui accompagnera les établissements sur les projets d'investissement les plus importants, en s'appuyant sur les recommandations d'un conseil scientifique et technique. Afin de permettre l'exercice d'une pleine démocratie sanitaire sur des décisions structurantes pour notre système de santé et pour nos territoires, il est proposé que le CNIS intègre des représentants des fédérations les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, ainsi que des représentants des usagers du système de santé et des élus locaux,

Le Gouvernement s'est engagé, à l'issue du Ségur de la santé, à mieux ancrer les politiques de santé dans les territoires et à associer davantage les élus locaux aux décisions d'investissement,

lequel a vocation à accompagner les établissements sur les projets d'investissements les plus importants et devrait offrir un cadre de pilotage intéressant et, de ce fait, une meilleure lisibilité en ce qui concerne, notamment, la répartition des ressources. Cet amendement vise donc à préciser dès à présent le rôle et la composition de cette nouvelle instance et à associer, aux représentants des services de l'État et des organismes nationaux de l'assurance maladie,

outre, les précisions apportées quant au fonctionnement du CNIS, sa composition et ses compétences, jusqu'aux modalités de traitement des demandes, excèdent largement ce qu'il est nécessaire d'inscrire dans le champ législatif. Je rappelle que le Copermo n'était pas prévu par la loi. Alors qu'une concertation est en cours et que les préoccupations soulevées par ces amendements sont satisfaites,

Il est proposé, pour s'assurer que celle-ci est saisie, qu'un rapport soit présenté au Parlement au 1 septembre 2021, recensant et détaillant les investissements dans les services hospitaliers situés dans les zones de revitalisation rurale

des crédits soient sanctuarisés pour ces territoires ruraux. Quel

Il avait alors estimé que cette dette, essentiellement immobilière et résultant de plans d'initiative gouvernementale, ne relevait pas de la dette sociale et, partant, n'avait pas à être amortie par la Cades. Le Gouvernement n'a cessé de soutenir sa position initiale au cours de la discussion parlementaire

nous estimons que les modalités retenues et traduites dans cet article ne sont pas toujours conformes aux exigences organiques. Il appartiendra au Conseil constitutionnel d'en juger. d'en juger. Ces modalités conduisant à faire financer par la Cades la reprise d'une dette des établissements de santé qui relève, par essence, de l'État, elles privent la sécurité sociale d'une ressource nécessaire à son équilibre financier. Ainsi la rédaction transmise par l'Assemblée nationale tend-elle à effacer le lien entre les dotations de la CNAM et les encours de dette des établissements au profit d'une mise en valeur de l'investissement. Le Gouvernement précise que la référence à des investissements futurs vise à garantir la conformité du dispositif à la réglementation européenne relative aux aides d'État, laquelle ne saurait admettre qu'une aide en vue d'investissements à venir.

Cela renforce la démarche qui nous a conduits à demander la suppression de ces dispositions. La présentation de cet article après le raisonnement soutenu cet été sur la loi relative à la dette sociale est donc toujours paradoxale et contribue, je le dis de nouveau, à transformer dans les faits la Cades en fonds d'investissement pour les hôpitaux, ce qu'elle n'a pas vocation à être.

d'intérêt collectif s'élève à 32 milliards d'euros en 2018. Ce sont 41 % des établissements qui se trouvent en situation d'endettement à la suite des plans Hôpital 2007 et 2012 et en raison des funestes emprunts toxiques. Nous en connaissons tous les conséquences : les investissements et les modernisations ont chuté dans de nombreux établissements, laissant des bâtiments en mauvais état, voire délabrés, et entraînant des manques de matériels et d'équipements pourtant indispensables pour les soignants. soignants. L'exemple de l'hôpital André-Grégoire de Montreuil est parlant. Le maire, mon ami Patrice Bessac, se bat depuis des mois pour faire annuler la totalité des 98 millions d'euros de dette qui pèsent sur le fonctionnement quotidien et sur l'attractivité de cet hôpital de Seine-Saint-Denis. Cet article 27 pose problème pour deux raisons supplémentaires. Non seulement le Gouvernement ne reprend qu'un tiers de la dette, ce qui est insuffisant, mais, comme l'a dit Corinne Imbert, il se défausse sur la Cades, ce que dénonce à juste titre l'ensemble de la commission. Pourquoi l'État n'a-t-il pas fait le choix de mobiliser des crédits supplémentaires, plutôt que d'alourdir une nouvelle fois les déficits sociaux ? De plus, cette reprise de la dette est conditionnée à la signature d'un contrat avec les ARS et nous craignons fortement que cette contractualisation ne serve de prétexte pour justifier de futures coupes budgétaires dans les établissements. On le voit, cette mesure n'améliorera ni la situation dans les établissements ni les conditions de travail des soignants, pas plus que la prise en charge des patients. C'est pourquoi nous soutenons cet amendement de suppression.

Mais il faut savoir également que les établissements sont contraints à des normes, à des exigences, à la certification, à l'accréditation. Tout cela nécessite des dépenses. Il faut des systèmes de pour certains équipements.

pour lesquels il y a des certificats d'exclusivité, que ce soit au niveau de la maintenance préventive ou au niveau de la maintenance curative. Les experts visiteurs qui viennent chez nous, dans les outre-mer, ne prennent pas un train ni leur voiture personnelle. Ils prennent l'avion et leur billet est payé par les établissements,

qui a comme mission de financer la dette cumulée du régime général de la sécurité sociale. Or l'essentiel de la dette hospitalière est lié à des investissements immobiliers et ne relève pas de dépenses d'assurance maladie. Je vous rappelle qu'il y a un an le Gouvernement avait présenté les contours d'un programme massif de reprise de dette de 10 milliards d'euros sur trois ans, soit plus de 3,3 milliards d'euros par an destinés à restaurer l'équilibre financier des établissements. Un projet de loi devait être présenté au premier semestre 2020 en même temps que la loi de programmation des finances publiques pour préciser les modalités de cette reprise. Mes chers collègues, il semblait à l'époque que c'était à l'État et non à la Cades d'opérer cette reprise. Aux termes de deux lois du 7 août 2020, l'intervention de la Cades était en effet en priorité dédiée au désendettement des hôpitaux afin d'éviter, selon l'étude d'impact, que le niveau d'endettement ne menace dans certains cas la pérennité de leur mission permanente de service public à laquelle ils ne peuvent se soustraire. La rédaction de l'article 27 tend pourtant à orienter davantage cette intervention vers le soutien à l'investissement et à la transformation de l'offre, en redonnant aux établissements des marges financières nécessaires.

les promesses qui avaient été faites l'année dernière et les engagements du Gouvernement pour rembourser la dette de l'hôpital ne m'avaient pas échappé puisque tout cela entrait en partie dans ma mission de contrôle de la dette. Nous nous posions la question,

mais une mesure de solidarité et de refinancement. C'est une mesure de solidarité, car elle vise à aider les établissements les plus fragilisés. C'est une mesure de refinancement, car elle permet aussi de s'appuyer sur des taux actuellement très bas. Les conditions de financement de la Cades sont en effet beaucoup plus favorables que pour les établissements de santé, surtout lorsque la durée d'amortissement est limitée. Le Gouvernement a fait évoluer la mesure initialement prévue pour la réorienter plus explicitement vers l'investissement, vers la transformation de l'offre du service public hospitalier.

que la Cades a été créée dans les années 1990 pour rembourser la dette sociale. Reprendre une partie de la dette immobilière des hôpitaux pour la transférer dans la dette sociale, c'est considérer, encore une fois, que l'immobilier des hôpitaux est une dette sociale.

et sociale, et pénalisera certains patients qui n'ont parfois pas d'autre choix que de consulter les urgences. Elle pourrait ainsi limiter l'accessibilité des soins aux personnes précaires dans un contexte d'aggravation des inégalités sociales et de santé.

est d'une complexité confondante. On parle de cet enjeu depuis plusieurs années et vous nous proposez une nouvelle expérimentation de cinq ans dont on peine à comprendre la mise en place concrète et les effets sur les finances des établissements. Comment sera déterminée la répartition entre la dotation socle et la part récente de tarification à l'activité (T2A) ? Quels critères présideront à la fixation des dotations socles ? Comment imaginez-vous l'évolution de cette dotation et celle de la T2A ? Quels critères présideront à la fixation de la dotation populationnelle ?

En outre, et j'en viens à mon amendement, nous ne trouvons rien dans ce PLFSS qui permettrait de travailler à une meilleure coordination entre la médecine de ville et l'hôpital. C'est pourtant un sujet dont nous discutons également depuis de nombreuses années. revanche, vous nous proposez encore une fois un dispositif de financement sur les urgences : pas de surprise, il y en a un à chaque PLFSS ! En 2019, nous avions eu droit au forfait de réorientation,

Madame la ministre, tout cela témoigne d'une façon d'aborder la question des urgences qui ne change rien ! C'est non par des mesures financières que l'on régulera

Je citerai Philippe Batifoulier, professeur d'université en santé et protection sociale : il estime que le nouveau forfait, comme la plupart des forfaits, est une aberration économique et pose un problème de santé publique. C'est une analyse que nous partageons. Déplorant que le nombre de passages annuels aux urgences ait doublé depuis vingt ans, le Gouvernement ne dresse pas de bilan de son incapacité à construire une offre de soins cohérente sur le territoire. Au contraire, il élabore une réforme visant à modifier le comportement des usagers en ce qui concerne le recours aux urgences,

le terrain. Étant donné les conditions d'accueil et les temps d'attente aux urgences, toujours plus catastrophiques en raison du manque de moyens criant des services et de la déficience des permanences de soins de la médecine de ville, comment peut-on voir un quelconque opportunisme des assurés dans

Pour rappel, 5 millions de personnes n'ont pas de complémentaire santé. On sait qu'aller se faire soigner est toujours une démarche difficile pour ces publics. Cette mesure ouvre donc la porte à des reports de soins qui,, engendreront des coûts importants pour la sécurité sociale. Elle ouvre aussi, bien évidemment, un nouveau marché aux complémentaires et constitue un pas de plus vers la marchandisation des soins. Une solution : le 100 % sécu pour tous et pour l'ensemble des soins

La simplification de la tarification des urgences par la création d'un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne saurait se traduire par un recul de droits pour les usagers. Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu'à présent inexistant, notamment pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l'affection longue durée (ALD) lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD, pour les donneurs en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits, ou encore pour les titulaires d'une pension d'invalidité.

révolter ! La régulation par l'argent en matière de santé, on connaît, hélas ! depuis un certain temps. Rappelez-vous, c'était en réduisant le nombre de médecins qu'on allait diminuer les dépenses ... Bilan des courses, on n'a plus de médecins ! Ici, on nous

La consultation de l'association France Assos Santé s'imposait également pour évaluer l'impact de cette mesure sur les inégalités de santé, le renoncement aux soins ou leurs reports. Le principe de forfaitisation n'est pas en cause. Les tickets modérateurs à l'acte, même plafonnés, comportaient le risque de leur multiplication non pertinente et donc de gaspillage. Le risque est bien celui la hausse régulière de ce type de forfait qui ne saurait participer d'un report plus grand des frais de santé sur les usagers, directement ou leurs mutuelles, qui se traduit par l'augmentation constante des tarifs. Cependant, en n'excluant pas de ce forfait tous les patients précédemment exonérés de ticket modérateur, pour lesquels est prévu un forfait réduit, cette modification participe à l'augmentation du reste à charge dans un contexte particulièrement inopportun de crise sanitaire et sociale. Cet amendement vise donc à maintenir leurs situations d'exonération en les excluant du paiement du forfait unique urgences, afin de ne pas altérer leurs accès aux soins. Quel que soit le dispositif, l'amélioration de l'accès aux droits et à la santé est une préoccupation constante du groupe écologiste, ce qui explique son soutien aux politiques de lutte contre le non-recours. Le modèle de financement des structures des urgences sera fondamentalement régulé par la réduction des causes du recours aux urgences pour des raisons sociales ou de carence de l'offre en ville, estimées à plus de 30 % par certains urgentistes. Cela nécessite une réforme ambitieuse de l'organisation des soins en ville et sur l'ensemble du territoire, réforme qui devrait s'accompagner, à défaut de la précéder, d'une réforme du financement.

les patients bénéficiaires du dispositif de l'ALD. Le remplacement du ticket modérateur par le « forfait patient urgences » semble créer un reste à charge jusqu'ici inexistant

du forfait. Cela revient à nier le principe même du régime de l'ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé. Les deux

en lieu et place du ticket modérateur pour le passage aux urgences non suivies d'une hospitalisation. Je partage le sentiment de perte de sens lié à des réformes par petites touches. Je souscris également au fait que le remplacement du ticket modérateur par une participation forfaitaire ne constitue pas une réforme structurelle pour les urgences hospitalières, comme l'a rappelé M. Jomier, sujet sur lequel nos collègues Laurence Cohen et René-Paul Savary ont travaillé de manière approfondie en 2017. Cette réforme, avant tout technique, représente toutefois une simplification pour les hôpitaux alors qu'aujourd'hui une part significative des factures n'est pas recouvrée. C'est aussi un gage de meilleure lisibilité pour les patients. ¨Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements. Les autres amendements Les autres amendements tendent, avec quelques nuances, à revenir sur le champ des exonérations à cette nouvelle participation forfaitaire « urgences ». Il s'agit de proposer l'exonération totale de forfait pour les personnes qui bénéficient à l'heure actuelle d'une exonération du ticket modérateur. L'Assemblée nationale a déjà engagé une évolution en ce sens concernant les femmes enceintes ou les nouveau-nés. Je comprends que l'intention du Gouvernement était d'instaurer une plus grande mutualisation puisque les personnes en ALD, quand elles vont aux urgences pour un problème sans lien avec cette affection, ont en général un reste à charge élevé. Celui-ci serait plafonné avec le principe de forfaitisation. Toutefois, la commission soutient, au nom d'une certaine équité, le maintien d'une exonération totale pour certaines catégories de patients aujourd'hui déjà exonérés, notamment ceux qui sont en ALD. En revanche, l'exonération pour les donneurs d'organes prévue par les amendements identiques

Par ailleurs, son montant est minoré pour les patients qui bénéficient d'un régime d'exonération. Deuxièmement, elle vise la lisibilité du coût des passages aux urgences et du montant du reste à charge des patients. Troisièmement, elle vise la simplification administrative, qui permet des gains de temps et de gestion pour les établissements. réclament ces simplifications afin de pouvoir se recentrer sur leurs missions essentielles, au profit de l'ensemble des patients. Enfin, je rappelle que 96 % des assurés disposent d'une couverture complémentaire. Cette participation forfaitaire sera également prise en charge.

un avis défavorable.

Or, vous le savez, cela n'aura aucun effet en la matière. Ces mesures sont vouées à l'échec. Le plus désolant, encore une fois, c'est que vous ne nous proposez aucune mesure structurelle

Nous avons, comme vous le savez, engagé une réforme en profondeur du mode de financement des établissements de santé. Il s'agit, notamment, de remplacer progressivement la tarification à l'activité par des modes de financement plus mixtes, qui tiennent davantage la pertinence et de la qualité des prises en charge. Si le Ségur de la santé nous a conduits à réaffirmer cet objectif, la deuxième vague de la covid-19 et la crise sanitaire que nous traversons nous obligent à reporter cette réforme.

à but lucratif. En effet, l'année 2020 a été fortement marquée par la lutte contre l'épidémie de covid-19, à tel point que toutes les catégories d'établissements de santé ont été mobilisées,

Pourtant, dans cette perspective de lutte prolongée contre l'épidémie, le projet de loi de financement de la sécurité sociale maintient la mise en oeuvre de la réforme du financement des activités de soins psychiatriques, dès le 1 janvier 2021. Une telle précipitation, en pleine période de gestion de crise sanitaire, n'apparaît ni raisonnable ni opportune, alors que nous

: La parole est à M. Martin Lévrier. La mise en oeuvre de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, prévue à partir de 2021, avec des mesures transitoires, s'effectuera par étapes.

En effet, les établissements qui bénéficient du prix de journée « tout compris » sont dans une situation tarifaire dérogatoire, car ils ne peuvent pas facturer d'honoraires médicaux. Pour rappel, ce régime dérogatoire a été mis en place dans certaines régions, sous l'impulsion des ARS. La moitié de ces établissements sont financés par un prix de journée qui couvre la rémunération de médecins salariés, avec une totale absence de facturation aux patients. L'autre moitié fait intervenir des médecins et auxiliaires médicaux libéraux dont les honoraires sont facturés en sus du prix de journée. Ce rattachement à la tarification des Espic admis à participer au service public hospitalier permet de simplifier les modes de financement des activités de soins de suite et de réadaptation, et de rétablir l'égalité tarifaire avec les autres catégories d'établissements de santé privés qui participent au service public hospitalier.

Je vous remercie

aussi, une nouvelle fois, d'un an le modèle transitoire de financement des activités de SSR, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Enfin, il reporte d'un an, à 2022, l'entrée en vigueur de la réforme du financement des activités de psychiatrie votée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

redoutent une standardisation des soins, une perte de temps à répondre à ces protocoles, au détriment du soin personnalisé qu'il faut apporter à chaque patient.

Quel est l'avis de la commission ? Le Sénat s'était opposé quasi unanimement à cette disposition lors de l'examen du PLFSS pour 2019, et la logique ne nous semble toujours pas vertueuse. L'arrêté du 27 décembre 2019 a fixé le cahier des charges de l'expérimentation

de ville et l'hôpital. Or l'expérimentation de forfaits repose, en premier lieu, sur un travail conjoint entre les urgentistes et les praticiens libéraux

Si le reste à charge qui est effectivement payé par le patient, après intervention des organismes complémentaires, demeure globalement faible à l'hôpital public, les montants sont très variables et peuvent être très élevés dans certaines situations.

De plus, ces restes à charge peuvent être très difficiles à supporter pour les patients qui n'ont pas de couverture complémentaire. Ce sont donc les patients les plus âgés, les plus malades et les plus démunis

en effet, que plus de 96 % des assurés ont signé un contrat de complémentaire santé responsable, qui couvre obligatoirement la participation de l'assuré aux frais liés à la prise en charge de l'hôpital. Ce contrat doit permettre aux assurés de bénéficier du tiers payant sur ces frais, à hauteur du ticket modérateur. conséquent, cet amendement comporte un risque financier réel pour l'assurance maladie, en cas de difficultés de recouvrement de cette avance de frais. Par ailleurs, je précise que pour tenir compte du contexte actuel, le Gouvernement a déposé un amendement visant à reporter d'un an l'entrée en vigueur de certaines réformes du financement des établissements de santé, prévues en 2021, dont la réforme du calcul du ticket modérateur. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement

de la commission ? Il est vrai que les règles sanitaires actuelles conduisent à privilégier la chambre individuelle pour les hospitalisations. Cependant l'amendement, tel qu'il est rédigé, ne me paraît pas répondre de manière satisfaisante au besoin de prise en charge de cette prestation, car il entraînerait une perte de recettes pour les établissements de santé.

qui est transmis au Parlement. De plus, un rapport sur le financement des établissements de santé, établi en application de l'article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale, présente en annexe la ventilation des missions

inutiles, en faisant de la pertinence des soins un sujet de discussion entre les ARS et les établissements, au même titre que l'efficience ou la qualité des soins, afin de réorienter les ressources vers les soins pertinents et les actions de prévention menées au sein des établissements de santé.

avec les acteurs locaux. Cet amendement tend à renforcer les dispositions existantes en donnant une portée financière systématique à tout manquement objectivé et répété aux critères de pertinence des soins.

La réforme du financement des activités d'urgences, de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation s'inscrit dans le cadre d'une régionalisation de l'allocation des ressources financières des activités de santé. La consolidation du rôle des ARS qui s'ensuit nécessite donc une plus grande transparence. C'est pourquoi le présent amendement vise à fixer dans la loi la nécessité, pour le directeur général de l'agence régionale de santé, d'informer la conférence régionale de la santé et de l'autonomie

nécessaires ? La transparence est cruciale pour toute politique publique. Aussi, cet amendement prévoit de donner les moyens à cette conférence d'être un acteur clé de la gouvernance de santé.

Un objectif unanimement partagé de simplification impérative des règles et des circuits de facturation a été posé et repris dans les conclusions du rapport de Mme Notat. Dans ce contexte, il paraît contradictoire, voire contre-productif, d'imposer aux établissements publics de santé, contre leur volonté, une facturation individuelle qui alourdirait et complexifierait de façon significative les tâches de facturation, et engendrerait des rejets à traiter et des retards de paiement.

Les préoccupations des auteurs de cette disposition quant au développement insuffisant, en France, de l'autodialyse ou de la dialyse à domicile sont légitimes ; à titre personnel, je les partage. Toutefois, le recours à l'une ou l'autre de ces pratiques relève d'abord du colloque singulier entre le médecin et son patient. De surcroît, la précision apportée ne relève pas du niveau législatif, puisque la puisque la définition des indicateurs est fixée par voie réglementaire. C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.

doit être un établissement doté d'un service d'urgences, d'une maternité de niveau 1, au minimum, et de services de médecine. Ces établissements doivent aussi avoir un service de soins de suite et une structure pour les personnes âgées. Enfin, ils doivent être un lien avec la médecine de ville et, éventuellement, avec les centres de santé et la psychiatrie de secteur. C'est ainsi, me semble-t-il, que nous pourrons redonner envie aux jeunes médecins de venir s'installer dans des territoires plus isolés et de travailler à l'hôpital public. Cet article est important, car il ne suffit pas d'élaborer de nouvelles dispositions encore faut-il en dresser le bilan, évaluer leur utilité ou leur nocivité. Il est essentiel, pour les parlementaires que nous sommes, de disposer d'une évaluation de la labellisation et du développement des hôpitaux de proximité. Aussi, tout en connaissant la position du Sénat sur les demandes de rapport,

L'état de vétusté de nos hôpitaux et leurs difficultés financières s'expliquent par les modalités de financement de nos hôpitaux publics, fondées sur la T2A, laquelle est totalement inadaptée à la prise en compte de la pertinence des soins

Ce n'est pas l'expérimentation du modèle mixte de financement des activités de médecine prévu à l'article 29 qui va redonner du souffle à nos hôpitaux publics. Répondre à une prise en charge globale a un coût. Celui-ci n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la ministre, de réponse structurelle de long terme au problème de financement des hôpitaux.

Je vous propose, par cet amendement que je présente au nom de la commission, de circonscrire le champ de cet article qui répond à une ambition louable, mais qui nous semble traduire une certaine impréparation. En effet, si nous partageons l'objectif d'une diversification des financements de l'hôpital, les contours du dispositif proposé sont, à ce stade, très imprécis. Je comprends que le Gouvernement entende poursuivre ses travaux. Un travail de coconstruction avec les acteurs concernés est évoqué. Cela est, bien entendu, nécessaire. Toutefois, rien n'est dit à ce stade sur le champ des activités concernées, la coopération avec le secteur ambulatoire ou encore l'articulation avec d'autres dispositifs sur lesquels nous n'avons pas encore de retour, comme le financement forfaitaire des pathologies chroniques voté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Or le contexte actuel me semble peu propice à l'incertitude sur le financement des établissements de santé. L'amendement vise donc à s'en tenir à la première étape envisagée, à savoir la dotation socle, opérationnelle dès 2021. Cela permettra d'offrir une option aux établissements volontaires, dont le premier bilan sera utile pour se prononcer, dans un prochain PLFSS, sur les contours plus précis de l'expérimentation et d'apprécier son potentiel impact financier. Cet amendement tend par ailleurs à introduire une évaluation sur la base, notamment, d'indicateurs liés à la pertinence et à la qualité des prises en charge, ainsi qu'à la coordination ville-hôpital-médico-social, critères essentiels, selon nous, à la prise en charge des pathologies chroniques ou des patients âgés.

entre régions. Elle doit aussi favoriser les coopérations à l'échelle du territoire, au service d'une meilleure pertinence des soins et de la prévention. À ce titre, cet amendement a pour objet d'étendre le périmètre de la dotation populationnelle aux activités de chirurgie et d'obstétrique

sur des objectifs de qualité des prises en charge et de réponse aux besoins du territoire tiendra bien compte de la nécessaire coordination ville-hôpital. En effet, dans certains territoires, cette coordination dans le domaine de la cancérologie était déjà fragile avant l'épidémie de covid-19. Les structures ambulatoires de soins curatifs et palliatifs étaient inégalement disponibles en fonction des lieux de vie des individus. Par conséquent, pendant cette période de crise, certains acteurs de terrain ont témoigné de situations très difficiles pour les personnes malades, contraintes d'être soignées à domicile : isolement extrême, interruption de certains soins pendant la période du confinement, gestion des soins palliatifs par les aidants et difficile coordination entre les services d'hospitalisation Afin de s'assurer que ce besoin de coordination essentiel aux territoires, et surtout aux personnes malades, sera pris en compte dans les conditions d'entrée dans le dispositif, le présent amendement tend à modifier l'article 29 pour y inclure l'objectif annoncé par le Gouvernement dans son exposé des motifs. ce besoin de coordination pourrait notamment s'apprécier au regard des moyens alloués par l'établissement à la création de postes d'infirmiers de coordination.

simple d'application de l'article 29. Ce montant sera fixé par arrêté, qui est le niveau réglementaire le plus adéquat. Par conséquent, le décret d'application précisera les modalités d'entrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, ainsi que les modalités de détermination et de calcul de la dotation socle. L'amendement n° à M. Alain Milon. Cet amendement vise à s'assurer que la contractualisation avec l'ARS sur des objectifs de qualité des prises en charge et de réponse aux besoins du territoire tiendra bien compte de la nécessaire coordination ville-hôpital, primordiale lorsqu'un lorsqu'un patient est atteint par la maladie du cancer.

Enfin, l'amendement de Mme Jasmin est effectivement satisfait. Les coefficients géographiques applicables aux établissements d'outre-mer s'appliquent aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels. Il semblerait normal que ce soit aussi le cas de la dotation socle.

Cet objectif, que nous partageons, est pris en compte dans les axes stratégiques du développement de l'HAD et décliné dans les travaux menés par les services du ministère concernant le financement des activités de soin. journées d'hospitalisation à domicile a augmenté de 7 % en 2019, après des années d'évolution positive. La réforme en cours du financement de l'HAD prévoit la mise en place d'un compartiment incitatif à la qualité.

» -sur la révision du coefficient géographique pour les établissements publics de santé ultramarins. En effet, le coefficient actuel n'est plus adapté aux réalités des coûts locaux. Pour La Réunion, par exemple, le coefficient a connu une augmentation d'un point en douze ans. de la commission ? Nous avons déjà prévu, à l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la remise d'un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l'article 73 de la Constitution

avait été portée par notre ancienne collègue centriste Muguette Dini. Une excellente collègue ! Au nombre de huit, ces lieux de suivi de grossesse et d'accouchement sont gérés

à nous émouvoir de la réponse tardive du Gouvernement quant à l'absence de visibilité subie par les huit maisons de naissance. La loi du 17 juin dernier a prolongé leur expérimentation d'un an.

Loin de se substituer aux maternités classiques, les maisons de naissance renforceront utilement le maillage sanitaire de nos territoires. Je tiens, pour terminer, à saluer le rôle des sages-femmes, qui sont impliquées à tous les niveaux de gestion et qui ont permis à chaque maison de naissance de s'adapter à son contexte local.

L'article 30 prévoit de pérenniser les maisons de naissance, structures autonomes de suivi de la grossesse, de l'accouchement et de ses suites, placées sous la responsabilité exclusive des sages-femmes, propices à la tenue d'actions de prévention et d'éducation thérapeutique. La pérennisation des maisons de naissance pourrait aussi être une opportunité de suivre les recommandations émises dans le rapport de Nicole Notat. Celle-ci préconisait d'amplifier « la diversification des stages en centres hospitaliers, en Ehpad, en maison de santé pluridisciplinaire, en libéral » pour les étudiants en médecine. Or, dans le cadre de leur formation, ceux-ci doivent assurer le suivi médical des grossesses physiologiques et les soins du post-partum. Ainsi, les maisons de naissance pourraient constituer des lieux de stage en vue de la formation des étudiants sages-femmes, mais aussi des étudiants en médecine de troisième cycle. Cette mutualisation des compétences favorisera, par ailleurs, un meilleur exercice interprofessionnel futur. Aussi, afin de tirer le plus grand profit de la pérennisation des maisons de naissance, l'amendement n° 884 rectifié vise à leur ajouter de nouvelles attributions en matière de prévention et d'accueil de stagiaires.

mais peinent à répondre à toutes les demandes, démontrant qu'elles représentent une diversification de l'offre de soins périnatale attendue par de nombreuses femmes qui souhaitent, en outre, accoucher dans un environnement différent. Afin de répondre à cette demande croissante, cet amendement tend à offrir aux étudiants et aux sages-femmes qui le demandent la possibilité de se former au sein de ces maisons de naissance, de manière à mieux appréhender les accouchements ainsi que la prise en charge globale des femmes. En effet, ces maisons de naissance constituent aujourd'hui les meilleurs lieux de stage pour se former à cette prise en charge recommandée par la Haute Autorité de santé

Vous proposez de compléter les missions des maisons de naissance. L'article 30, tel qu'il vous est soumis, définit avec clarté ce qui fait l'essence même des maisons de naissance : le suivi de la grossesse et la réalisation des accouchements. Néanmoins, l'expérimentation qui a été menée ces dernières années et qui a fait l'objet d'évaluations a montré que, au-delà de ce socle de missions, d'autres approches pouvaient et devaient être développées par les maisons de naissance, comme le suivi postnatal ou le soutien à la parentalité. Je suis convaincue que c'est l'un des atouts de ce modèle qui va venir compléter l'offre en place. Ne pas mentionner dans le texte législatif d'autres missions, telles que la prévention ou l'éducation, n'empêchera pas leur réalisation par les sages-femmes et autres professionnels qui exerceront dans ces maisons, dans la mesure où ces missions font partie de leur champ de compétences. Cette possibilité étant préservée,

en permettant une juste tarification de la prestation de suivi et d'accompagnement global, ce qui rejoint les demandes des sages-femmes et de leurs syndicats : reconnaissance des astreintes du dernier mois, de la surveillance du travail d'accouchement, du immédiat,

choix de la contraception, choix du suivi pendant la grossesse, choix du type d'accouchement ... Si des femmes souhaitent effectuer un accouchement physiologique

Cet amendement vise à sécuriser la place et le rôle des sages-femmes au sein des maisons de naissance dont elles ont la charge. Depuis cinq ans, c'est-à-dire depuis le début de l'expérimentation prévue par la loi du 6 décembre 2013, la gestion médicale, technique, administrative et financière de ces structures a été assurée exclusivement par des sages-femmes, dans le respect strict du cahier des charges de la Haute Autorité de santé.

À l'Assemblée nationale, en première lecture, un amendement du rapporteur général de la commission des affaires sociales est venu préciser que la direction médicale de ces maisons était bien confiée aux seules sages-femmes.

en concertation avec les associations qui gèrent les huit maisons de naissance actuellement, de limiter le champ des organismes pouvant créer et gérer des maisons de naissance à des organismes à but non lucratif. Ce n'est donc pas tant la question du secteur public

l'amendement n° 397. Contrairement aux GCS, les GIE et les GIP ne peuvent pas porter une autorisation d'activité de soins et ne constituent pas des formes de coopération adaptées à l'objet même des maisons de naissance ou aux acteurs qui y participent. Cet amendement vise donc à retirer

la direction médicale des maisons de naissance par des sages-femmes est déjà réaffirmée dans le texte, ce qui confirme l'orientation prise dans le cadre de l'expérimentation. Faut-il ne confier leur gestion qu'à des sages-femmes ? Peut-être est-ce restrictif pour envisager le développement de ces structures

, visent à restreindre le type de structures susceptibles de créer et de gérer des maisons de naissance. Dès lors que le rôle central des sages-femmes dans ces structures me semble déjà garanti, je ne vois pas d'obstacle à élargir les possibilités de coopération pour faciliter le montage des projets, ne serait-ce que pour des questions de locaux ou de financement. Le cadre purement associatif des maisons de naissance a présenté

sur l'activité des maisons de naissance pourtant indispensable à leur suivi et à leur évaluation. Ce sont plus les conditions d'implantation des maisons de naissance qui importeront pour prévenir les effets de concurrence.

Toutes les données scientifiques dont nous avons connaissance sont positives quant à la qualité des soins en maison de naissance, sans qu'il y ait forcément une obligation de contiguïté. Le taux de transfert évoqué dans le débat parlementaire porte essentiellement sur des transferts non urgents. Comme l'explique l'étude de l'Inserm, les urgences majeures sont celles qui relèvent de l'hémorragie du. Pour Pour l'année 2018 sur laquelle porte cette étude, on relève ainsi 31 transferts en, soit 6 % des accouchements, généralement à la suite d'une hémorragie de la délivrance ou d'une rétention du placenta. Dans le premier cas, les gestes suffisants ont toujours été effectués par la sage-femme, et il n'est à déplorer aucun cas d'hospitalisation en unité de soins intensifs ou de réanimation. C'est donc non pas la contiguïté, mais le travail des sages-femmes et la qualité du partenariat et de la communication avec la maternité partenaire qui assurent le bon niveau de sécurité. La condition prévue par le texte actuel d'une convention « prévoyant, notamment, les modalités d'un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité paraît donc nécessaire et suffisante, sachant que les modalités pratiques permettant d'assurer ce transfert rapide seront cadrées dans les textes réglementaires s'appuyant sur le cahier des charges de la HAS et sachant que les ARS seront attentives sur ce point lors de l'instruction des demandes et lors du contrôle des maisons de naissance.

afin, notamment, d'assouplir le critère de contiguïté des maisons de naissance à un établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique, en le remplaçant par les termes « proximité immédiate ». Or une telle modification est porteuse de risque en cas de complication périnatale. Le rapporteur général de l'Assemblée nationale l'a souligné lors des débats, en indiquant que le critère de la contiguïté est essentiel. En effet, il ressort de l'expérimentation menée depuis 2013 que les transferts d'une maison de naissance vers une maternité concernent en moyenne 22 % des accouchements durant le travail, sans parler des transferts postnataux. La loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance avait bien pris en compte ce risque, en prévoyant que la maison de naissance soit attenante à un établissement de soins. La contiguïté à une maternité disposant d'un plateau technique pouvant gérer les complications éventuelles est indispensable. Mon expérience de pédiatre de maternité me ramène aux années quatre-vingt : nous étions alors obligés d'aller chercher les nouveau-nés dans plusieurs petites maternités à proximité des

J'avoue que l'affaire est délicate, puisqu'il s'agit de trouver un équilibre entre libre-choix, sécurité et

notamment dans des situations où le transfert, même rapide, n'est pas possible pour la santé de la femme ou du nouveau-né. Cependant, il me semble plus sage, dans un premier temps, de maintenir cette exigence. Je rappelle que le taux de transfert en cours d'accouchement est assez élevé, de l'ordre de 22 %.

l'avis du Gouvernement ? des maisons de naissance assurant la sécurité des soins dispensés aux parturientes et aux nouveau-nés. Au-delà des situations d'hémorragie du que vous avez évoquées et qui composent la majeure partie des urgences maternelles, on ne peut écarter d'autres situations graves pour la mère, comme pour le nouveau-né, qui justifient une proximité immédiate avec la maternité. À l'occasion des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a accepté de passer de la notion de

par les établissements hospitaliers. Il faut tout de même avoir en tête que la création d'une maison de naissance, avec l'exigence bien normale de l'adossement sur une maternité,

Il faut donc entendre les réserves qui peuvent s'exprimer et prendre en compte le fait que la proximité immédiate est demandée, y compris

de la commission ? Depuis 2017, les bénéficiaires de l'assurance maternité bénéficient déjà du tiers payant pour la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.

? Les actes réalisés pour la prise en charge des femmes enceintes relevant de l'assurance maternité à compter du sixième mois sont d'ores et déjà dans le champ du tiers payant obligatoire, qu'il soit réalisé en maison de naissance ou non. Le Gouvernement est donc Cet amendement vise à donner plus de visibilité aux gestionnaires des maisons de naissances, en allongeant la période d'autorisation d'une année, ce qui correspond à mon avis au temps d'un retour sur investissement et de l'amortissement des investissements.

l'ensemble de la prise en charge d'un état de santé ou d'une maladie. Elles devraient se limiter aux points d'amélioration de cette prise en charge, identifiés à l'aide d'études de pratiques ou, en l'absence de telles études, à l'aide des avis et de l'expérience des professionnels de santé concernés par le thème.

Quel est l'avis du Gouvernement ? La mention de l'opposabilité des recommandations de la HAS relatives aux maisons de naissance, en particulier du cahier des charges qui leur est directement applicable, doit être préservée. Pour cette raison, je suis défavorable à cet amendement.

Mon amendement tend à préciser que le décret en Conseil d'État doit prendre en compte les conditions de prise en charge par l'assurance maladie de la rémunération des professionnels exerçant dans les maisons de naissance, à savoir les sages-femmes. En effet, si l'objectif du Gouvernement est non seulement de pérenniser, mais aussi de promouvoir le développement de ces structures essentielles à la diversification de l'offre périnatale et au choix des femmes, il est essentiel de prévoir au plus vite les modalités de leur financement pérenne. Cela passe notamment par la reconnaissance du travail des sages-femmes en maison de naissance, donc par la définition de la rémunération de leurs actes. Quel

est l'avis du Gouvernement ? Il est prévu de déléguer à ces structures des financements complémentaires, par l'intermédiaire du fonds d'intervention régional. Nous prenons en compte le fait que le financement par l'assurance maladie des actes réalisés par les professionnels ne suffit pas pour assurer l'équilibre économique des maisons de naissance, en raison du poids de certaines dépenses. Un tel dispositif ne remet pas en question, bien au contraire,

sages-femmes, à l'occasion du suivi des grossesses ou du suivi gynécologique et de contraception, sont amenées à prescrire des examens, afin, entre autres choses, de dépister d'éventuelles situations pathologiques. À ce titre, l'article L. 4151-4 du code de la santé publique prévoit que les sages-femmes peuvent prescrire tous les « examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession Or la réforme de l'assurance maladie du 13 août 2004 a instauré un dispositif reposant sur le choix, par chaque assuré ou ayant droit de 16 ans ou plus, d'un médecin traitant dans le cadre d'un parcours de soins coordonnés. Ce dispositif, louable dans son principe, a totalement oublié les sages-femmes dans le dispositif de suivi normal et banal des femmes. Ces dernières ne doivent pas être pénalisées lorsqu'elles sont orientées par une sage-femme vers un médecin spécialiste. Les sages-femmes doivent pouvoir exercer dans le respect des recommandations professionnelles et de leurs obligations législatives et déontologiques. L'obligation d'adresser à un médecin en cas de situation pathologique ne concerne pas uniquement le médecin gynécologue ou généraliste. Cette situation va dans le sens d'une altération du parcours de soins des femmes enceintes et à une non-économie pour les finances de la sécurité sociale. La reconnaissance des sages-femmes dans le cadre du parcours de soins coordonnés s'inscrirait également dans une démarche de maîtrise les dépenses de santé.

ne s'applique pas si le patient est adressé vers le médecin traitant par une sage-femme. Je ne sais pas si cette précision est utile, dans la mesure où certaines spécialités, notamment la gynécologie, sont déjà en accès direct, sans passer au préalable par le médecin traitant. Pour les

À l'instar des maisons de naissance, dont nous venons de parler, ou de la proposition d'expérimenter l'orientation des patients en amont des urgences par le biais de la téléconsultation, l'article 31 vise à désengorger l'hôpital et à le recentrer sur sa mission de soins médicaux. de poursuivre le travail amorcé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, qui a lancé l'expérimentation des hôtels hospitaliers. Ce sont 41 sites d'établissements de tous statuts, répartis sur l'ensemble du territoire national, qui ont participé à l'expérimentation dans le cadre d'un appel à projets national. Les résultats transmis semblent bien répondre aux objectifs et aux enjeux de l'expérimentation. Les hébergements non médicalisés ont bien bénéficié aux patients éloignés géographiquement, dans le cadre de prise en charge en ambulatoire, pour

Aussi l'article 31 tend-il à renforcer le soutien au développement des hôtels hospitaliers, pour rendre ce dispositif plus attractif pour le plus grand nombre d'établissements de santé et plus accessible pour les patients le souhaitant, ce dont je me réjouis. La montée en puissance du dispositif permettra également de mieux définir son modèle médico-économique à long terme. Je souhaite cependant appeler l'attention de Mme la ministre, sur le cas de patients en situation de handicap ou en perte d'autonomie, qui ont besoin d'être accompagnés par un aidant pour accomplir leurs démarches. Dans la perspective d'une société plus inclusive et d'une reconnaissance du rôle crucial des proches aidants, je sollicite votre avis, madame la ministre, sur l'ouverture aux aidants familiaux de l'accès aux hôtels hospitaliers sans reste à charge.

Ces structures d'hébergement non médicalisées portent l'ambition de réduire les durées d'hospitalisation, en permettant un séjour avant ou après une intervention programmée à l'hôpital. Ces hôtels hospitaliers sont un appui à la médecine ambulatoire et répondent à la composition de la carte sanitaire. Si, dorénavant, ce ne sont pas dans les hôpitaux locaux que certains soins sont prodigués, les patients devront se déplacer plus loin, parfois le jour même de leur hospitalisation. Il est donc essentiel de pouvoir compter sur des solutions d'hébergement à proximité des hôpitaux. Le CHU de Nantes dispose d'ailleurs déjà d'une maison hospitalière, gérée par une association délégataire. On peut aisément penser que les nuitées assurées dans ces hôtels permettront de mieux utiliser les chambres hospitalières et de maîtriser les dépenses de santé. Toutefois, si nous sommes favorables au développement de ces structures, il nous a semblé nécessaire d'apporter quelques garanties qui concerne les usagères et les usagers les plus précaires. Ainsi, nous ne pourrions soutenir le recours accru à ces hôtels, s'il s'avérait qu'il introduit une augmentation du reste à charge par rapport à l'hospitalisation classique. Faute d'avoir été considéré comme recevable, notre amendement visant à permettre la prise en charge du coût de l'hôtellerie hospitalière pour les plus précaires ne pourra pas être examiné. En revanche, nous proposerons, par un autre amendement, que soit évalué le montant de ce reste à charge, notamment pour le public précaire ou isolé.

Bien souvent, les patients restent des heures sur les brancards. Ensuite, la saturation des hôpitaux permet de justifier un confinement total de la population, comme nous l'avons vécu au printemps dernier, et comme nous sommes en train de le vivre. Telle est la réalité ! Alors je ne peux m'empêcher de penser que ces hôtels hospitaliers sont une façon d'externaliser nos capacités hospitalières et de les privatiser. Par ailleurs, je m'interroge sur la pertinence de cette généralisation. Alors que l'objectif quantitatif de ces hôtels hospitaliers avait été fixé à 35 000 séjours et 56 000 nuitées d'hébergement non médicalisées, les résultats sont nettement en deçà, avec seulement 7 800 séjours et 17 500 nuitées, d'après l'annexe 9 du PLFSS. Bien sûr, j'entends l'argument relatif à la montée en puissance de ce dispositif encore trop méconnu, ainsi que celui sur la satisfaction des patients. Mais quand je constate que les questions de financement ne sont pas réglées, je m'interroge vraiment sur l'aspect prématuré d'une telle généralisation et sur sa dangerosité. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

le précise, le Gouvernement a engagé des travaux avec les fédérations hospitalières pour proposer un accompagnement financier suffisant permettant aux établissements de déployer les hôtels hospitaliers de façon soutenable. La commission soutient la généralisation de ce dispositif. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement. Quel

en assurant, pour les patients résidant loin des structures de soins, un accès aux services hospitaliers quand ils en ont besoin. Nous souhaitons généraliser le dispositif des hébergements temporaires non médicalisés, dont l'expérimentation a démontré les bénéfices en termes d'accès aux soins.

L'alinéa 3 de cet article permet à un hôpital de sous-traiter à un acteur privé la mise en place d'un dispositif d'hébergement non médicalisé pour les soins ambulatoires. Dans un contexte où les établissements de santé ont du mal à assumer leurs dépenses de fonctionnement, cela ouvre la voie à une privatisation rampante du service hospitalier. Cette mesure s'inscrit également dans la poursuite du virage ambulatoire, à l'origine de la fermeture, dans les hôpitaux, de lits dont nous manquons aujourd'hui pour faire face à la crise sanitaire. Or le développement des hôtels hospitaliers procède de la même logique, par l'externalisation de capacités hospitalières. Il s'agit en effet de continuer à remplacer les hospitalisations par des séjours en hôtels non médicalisés, afin de réaliser des économies. Il faut cesser de penser que l'hôpital est une compilation de services que l'on peut décider de privatiser lorsqu'il ne s'agit pas directement de soins. En réalité, l'hébergement est une composante du soin, car l'hôpital est un tout. Si la qualité des chambres d'hospitalisation est bien moindre à l'hôpital public que dans les hôtels hospitaliers, c'est en raison du désinvestissement financier de l'État depuis de

? Ma chère collègue, votre amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à un tiers pour externaliser la prestation d'hébergement hôtelier hors de l'établissement de santé. Or c'est le principe même de l'hôtel hospitalier : offrir la possibilité aux établissements de santé d'externaliser l'hébergement de patients ne nécessitant pas de prise en charge médicalisée, afin de mieux organiser les parcours de soins. J'ai rappelé précédemment l'intérêt de ce dispositif pour les patients et pour les établissements. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

pour ces territoires. Au fond, l'hôtel hospitalier, c'est la langue d'Ésope : la meilleure et la pire des choses. C'est la pire des choses si on le conçoit uniquement comme une source d'économies et de réduction de la durée des séjours hospitaliers. hospitaliers. C'est la meilleure des choses, en revanche, s'il représente une transition et une coordination entre la ville et l'hôpital, donc s'il permet, quand c'est possible, de réduire la durée de séjour, parce que personne n'a envie de rester à l'hôpital plus longtemps que nécessaire,

des transports sanitaires.

Vous indiquez d'ailleurs, dans l'objet de votre amendement, que ces entreprises de transport de personnes à mobilité réduite sont déjà soumises à des conventions avec la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Par conséquent, il ne m'apparaît pas opportun de créer dans la loi

allons parler, à l'article 32, des téléconsultations. La mise en place de la télémédecine ne date pas du confinement. L'assurance maladie en rembourse les actes depuis 2018, au même titre qu'une consultation en cabinet médical, avec ticket modérateur de 30 % pris en charge par les complémentaires. c'est bien le confinement qui en a permis l'essor. Ainsi, entre février et avril, le nombre de téléconsultations a été multiplié par plus de cent. Lors du premier confinement, ces actes ont été pris en charge intégralement par la sécurité sociale. C'est probablement le confinement plus que la prise en charge intégrale qui aura permis cet essor, n'en doutons pas. L'évidence est là : la téléconsultation fait désormais partie des nouvelles pratiques médicales. s'il faut s'en réjouir, la télémédecine ne doit pas devenir l'alpha et l'oméga du suivi de santé de demain. En effet, le meilleur écran et la meilleure « appli » qui soient ne remplaceront jamais le contact humain, lorsque de mauvais résultats d'analyse doivent être annoncés, par exemple. De même, une bonne télémédecine doit venir compléter la médecine « palpatrice », de chair et d'os, qui constitue la base du soin pratiqué par le médecin traitant, et doit s'insérer dans le cadre du parcours coordonné de soins. La téléconsultation est aussi un allié des territoires, à condition que les infrastructures numériques soient déployées. Elle peut pallier l'absence de médecins de campagne, et elle permet à tout patient d'avoir recours à la téléexpertise médicale sans avoir à se déplacer. Enfin, dernière réserve, n'oublions pas qu'un fossé numérique éloigne bon nombre de patients et de patientes du recours à cette médecine. Le Défenseur des droits nous a alertés sur les 13 millions de nos concitoyens qui ne maîtrisent pas les usages numériques. Envoi de documents, forfait téléphonique avec data : restons attentifs à ce qui permet ces consultations et levons les éventuels freins. Je soutiendrai donc l'initiative présentée par notre rapporteure visant à limiter la prise en charge intégrale aux téléconsultations réalisées dans le parcours de soins, avec une exception pour les consultations rendues nécessaires par la covid-19, qui doivent, elles, être intégralement remboursées, même hors parcours.

dans une moindre mesure, des consultations nécessaires aux parcours de soins classiques ou au suivi des maladies chroniques. Tout prête à croire- cela a été dit -que l'essor de la téléconsultation, à l'usage et l'expérience aidant, sera durable. La mesure proposée, à savoir la prise en charge à 100 % des téléconsultations indépendamment de leur nature, ne nous semble cependant pas Elle revient à considérer que cette forme de consultation pourrait se soustraire à la logique du parcours de soins, qui responsabilise le patient en l'invitant à des pratiques vertueuses. Ainsi le parcours de soins coordonné incite-t-il financièrement les patients à éviter le nomadisme médical et à ne pas multiplier les téléconsultations pour une même pathologie.

Au contraire, la dématérialisation inhérente à ce type de consultations, possibles depuis chez soi et par le biais de plusieurs opérateurs différents, peut inciter le patient à multiplier les téléconsultations, notamment pour se rassurer sur le diagnostic proposé. Il est donc nécessaire de considérer que la téléconsultation est une consultation à part entière, qu'elle a toute sa place dans le parcours de soins et que, en conséquence, elle est soumise aux mêmes règles de responsabilisation des patients. Tel est l'objet de cet amendement, qui vise à rappeler que la participation de l'assuré est liée au respect du parcours de soins et à préciser que les téléconsultations en lien avec la covid-19 sont intégralement prises en charge par la sécurité sociale. L'amendement

adaptée à l'incertitude sanitaire, qui se poursuit. Nous devons favoriser le recours à la téléconsultation pour ne pas retarder des diagnostics ni reporter des soins. Cependant, tel qu'il est rédigé, cet article manque d'encadrement ; son application pourrait conduire à des pratiques dégradées de la téléconsultation, éloignées du dialogue habituel entre les patients et leurs médecins traitants. C'est la raison pour laquelle le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose, cet amendement, que cette prise en charge à 100 % ne soit accordée qu'aux actes de consultation intervenant dans le cadre du parcours de soins coordonné. Cet encadrement, nous le motivons essentiellement par un souci d'égalité de traitement avec les consultations effectuées en cabinet. Il convient en outre de conserver les garde-fous que les parcours de soins instaurent contre certains comportements marginaux- tendance au nomadisme médical ou à la multiplication des consultations -, qui ne sont pas souhaitables pour la maîtrise des dépenses de santé. En revanche, compte tenu du contexte pandémique lié à la covid-19, notre groupe précise que les téléconsultations effectuées hors parcours de soins, mais en rapport l'épidémie seront, elles, bien prises en charge à 100 %. Mme la rapporteure. Cet amendement vise, d'une part, à réduire la durée de la prise en charge à 100 % des téléconsultations à six mois au lieu d'un an, afin d'en réexaminer l'utilité selon l'évolution de la situation sanitaire, part, à s'assurer du lien essentiel à préserver avec la logique du parcours de soins, afin de garantir la qualité de la pratique, dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées. J'ajoute, comme je l'ai indiqué en commission, que j'ai rectifié l'amendement pour prendre en compte explicitement explicitement les actes liés à la covid-19, puisque c'est le contexte sanitaire qui justifie cette mesure dérogatoire. La téléconsultation, quel que soit son intérêt, notamment dans le contexte sanitaire actuel, ne peut remplacer le contact physique intrinsèque à l'exercice de la médecine- notre collègue Mme Meunier vient de le rappeler. La prise en charge à 100 % répond par ailleurs davantage à un objectif pratique qu'à une logique de santé publique : alors que cette mesure résulte d'un déploiement insuffisant des outils permettant la facturation des actes à distance, l'étude d'impact ne s'appuie sur aucune perspective

Une telle possibilité constituerait une dérogation aux conditions conventionnelles, qui prévoient que la prise en charge à 100 % par l'assurance maladie est conditionnée notamment au respect du parcours de soins, pour les consultations comme pour les téléconsultations. En l'état, l'article fait ainsi peser un risque important de dérégulation du secteur de la téléconsultation et d'augmentation des dépenses de santé afférentes. En effet, la prise en charge à 100 % de l'ensemble des téléconsultations par l'assurance maladie risque d'entraîner une déresponsabilisation des patients, ainsi que le développement de pratiques opportunistes de la part de certains professionnels de santé. Par ailleurs, elle aura pour effet de fragiliser le modèle économique des acteurs de la téléconsultation, qui ont avant tout besoin d'un cadre réglementaire et financier stable.

L'article 32 du présent PLFSS ne déroge pas aux conditions conventionnelles de réalisation et de prise en charge des téléconsultations. Le respect du parcours de soins coordonné est l'une des conditions fixées par les conventions.

peuvent être prises en charge à 100 % jusqu'au 31 décembre 2020, même si le parcours de soins coordonné n'est pas respecté. Cette dérogation prévue par décret pourra bien sûr être prolongée en fonction de l'évolution du contexte sanitaire. Je partage votre vision de la téléconsultation. Elle a rendu de grands services pendant cette crise sanitaire, notamment sur les territoires touchés par la désertification médicale. Pour autant, le lien humain doit être préservé. Tel est bien le sens de cet article 32, qui, donc, n'est pas

Les conditions de prise en charge de la téléconsultation sont définies par l'avenant n° 6 à la convention médicale : ces actes sont rémunérés à hauteur des tarifs des consultations en présentiel. Si je comprends et partage la volonté de mieux encadrer la prise en charge dérogatoire des téléconsultations

sanitaire, elle ne doit pas se substituer aux consultations en présentiel. Nous tenons à alerter sur le fait que la dématérialisation de la consultation médicale altère- pour le moins, transforme -le contact humain entre les praticiens et les patients. Ces rapports sont primordiaux : ils ne peuvent être remplacés par la technologie. De plus, certains examens médicaux ne peuvent pas être réalisés à distance. Alors que, pour être efficace, la télémédecine doit rester complémentaire d'un vrai suivi médical,

D'aucuns rêvent d'une société sans contact, qui limiterait les relations, tant individuelles que collectives, y compris dans les services publics ... Cet amendement vise à poursuivre l'utilisation de la télémédecine, sans la généraliser.

d'ailleurs ce qui a conduit le Gouvernement à y déroger face à l'épidémie de covid-19, en autorisant la consultation par téléphone dans certaines situations, notamment pour des patients âgés. Je ne vois pas d'obstacle à prolonger ces modalités dans les cas peu nombreux visés par les amendements. La commission Défavorable.

elle se révèle insuffisante pour la psychiatrie, spécialité durablement sinistrée. En effet, la prise en charge à 100 % ne dispense pas le patient de respecter le parcours de soins, notamment le critère de territorialité, pour être remboursé de sa téléconsultation.

dérogatoire à la logique de l'organisation territoriale. Je puis témoigner que, dans les situations de détresse dont je parle, une téléconsultation peut permettre de suivre avec un malade son évolution

Si le projet de numéro unique prévu dans le cadre du service d'accès aux soins contribuera à la bonne orientation d'une partie des patients, il ne pourra pas éviter les nombreuses arrivées directes de patients au sein des services d'urgence. À ce titre, la téléconsultation offre l'occasion de faciliter le triage des patients au sein même des établissements de santé disposant de services d'urgence. Les infirmiers organisateurs de l'accueil pourraient ainsi disposer d'une salle permettant d'effectuer les téléconsultations, afin d'orienter les patients, le cas échéant, vers une offre en de médecine ambulatoire. Les téléconsultations seraient assurées par des médecins du territoire, assurer ce type de prise en charge, renforcés en tant que de besoins par des médecins organisés au sein de plateformes de téléconsultation, en mesure de libérer le temps médical nécessaire à une prise en charge vingt-quatre heures sur Ces prises en charge devront bien sûr être enregistrées au sein du dossier médical partagé du patient. Aujourd'hui, le développement de services ou d'expérimentations d'une solution d'orientation des patients aux entrées des urgences par le biais d'un espace attenant de téléconsultation est freiné par le mode de rémunération de l'hôpital. En effet, ce service attenant, faisant intervenir du personnel hospitalier pour accueillir et orienter les patients et recourant à une plateforme de téléconsultation opérationnelle vingt-quatre heures sur ne peut être financé ni par l'hôpital ni par le patient. Cette innovation organisationnelle destinée à fluidifier les urgences doit s'accompagner d'une innovation structurelle et d'un financement spécifique. Pour impulser une volonté et une action collectives en faveur d'un tel dispositif, il est nécessaire d'identifier et de valoriser de façon objective les apports de la téléconsultation au sein des services d'accueil d'urgences, pour la santé publique comme pour les comptes publics. La parole est à M.

avis défavorable sur ces amendements

Ces étapes encouragent et soutiennent financièrement le déploiement de projets de télémédecine sur l'ensemble du territoire. La loi prévoit qu'un rapport d'évaluation pour l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé sera remis à la fin du mois de juin 2021,

de la commission ? L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a maintenu les actions de télésurveillance dans un cadre expérimental pour quatre ans, soit jusqu'en 2022, alors que la téléconsultation et la téléexpertise entraient dans le droit commun.

en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l'expérimentation.

de deux amendements identiques. utilisables par les opticiens-lunetiers et les orthoptistes en autonomie, sous le contrôle des ophtalmologistes, et l'élargissement de la téléexpertise aux relations entre ophtalmologistes et orthoptistes ou opticiens-lunetiers. préconisait de lancer une réflexion avec les professionnels de la filière sur la façon dont les nouveaux outils pourraient faire évoluer les stratégies de téléexpertise et de dépistage, ainsi que sur l'utilisation des réseaux en place, en particulier celui des opticiens-lunetiers.

entre les médecins et l'assurance maladie détermine les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins. L'adoption de cette disposition a été obtenue de haute lutte par le Sénat,

Cette mesure constitue une solution de substitution à la mise en place d'une régulation de l'installation des médecins par le conventionnement, qu'appellent de leurs voeux nombre de parlementaires et d'associations de patients et même la Cour des comptes, face à l'aggravation particulièrement préoccupante des déserts médicaux dans nos territoires,

La situation dramatique de nos territoires en matière d'accès aux soins n'autorise pas de repousser à plus tard cette négociation, comme le propose le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. C'est pourquoi cet amendement vise à

est très compliqué de faire une convention médicale juste avant une élection présidentielle, parce que, forcément, il y a des mécontents ... comme s'il ne suffisait pas que le rythme politique de notre pays soit entièrement réglé sur l'élection présidentielle, au point que notre démocratie parlementaire est singulièrement affaiblie, voilà maintenant que la démocratie sociale doit aussi être subordonnée à l'élection présidentielle

Les conclusions du Ségur de la santé, dans son volet ambulatoire, ont engagé d'importantes évolutions de l'activité des professionnels de santé libéraux. En conséquence, les partenaires conventionnels ont été invités à ouvrir des négociations autour des priorités issues du Ségur de la santé, notamment l'accès aux soins non programmés et le renforcement de l'exercice coordonné. Dans le contexte sanitaire actuel, le service d'accès aux soins, le SAS, qui doit permettre de soulager les services d'urgence, de même que le financement d'une nouvelle mission dédiée à la réponse aux crises sanitaires graves des communautés professionnelles territoriales de santé doivent être activés au plus tôt. Cela nécessite que les mesures conventionnelles qui doivent permettre leur déploiement soient mises en place au plus tôt en 2021. Or l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement que toute mesure conventionnelle ayant un impact financier ne peut entrer en vigueur qu'après un délai de six mois après son approbation. Au vu des enjeux essentiels portés par ces négociations, il convient de lever cette règle pour rendre d'application immédiate les modalités qui seront déclinées dans les conventions, de manière à garantir une montée en charge rapide de ces dispositifs sur le terrain. Cette dérogation à la règle habituelle permettra aussi une mise en oeuvre rapide des mesures conventionnelles actuellement négociées entre les entreprises de transport sanitaire et l'assurance maladie, qui permettront de mettre en oeuvre une réforme importante de la garde ambulancière, maillon essentiel de la réponse à l'urgence préhospitalière.

L. 162-1-9-1 prévoit la procédure de fixation des tarifs et de la classification des équipements matériels lourds, et la nature de l'avis, non conforme, de la commission. Il précise que le directeur général de l'Uncam transmet cet avis aux syndicats médicaux représentatifs, ainsi qu'au ministre de la santé. Faute d'accord avec les syndicats représentatifs, le directeur général fixe unilatéralement les tarifs et la classification des équipements lourds. Ces deux articles rompent avec les principes de la négociation conventionnelle et les procédures de fixation des tarifs qui en découlent. Sous couvert d'une concertation entre le entre le directeur général de l'Uncam, les professionnels et les établissements opérant un scanner, une IRM ou un TEP-scan, ainsi qu'avec les syndicats conventionnels, ils confèrent un pouvoir unilatéral

identiques visent à supprimer la commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale créée auprès de l'Uncam en 2017, commission qui détermine par une procédure spécifique les forfaits de radiologie. Lors de l'examen du PLFSS pour 2017,

du Gouvernement ? Cette disposition faisait suite à un rapport de la Cour des comptes de 2016, qui mettait en lumière l'inadéquation du mode de tarification de l'imagerie et les très forts effets de rente qui en découlaient, représentant des coûts de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros pour l'assurance maladie obligatoire.

Aussi la prise en charge à 100 % sans avance de frais représente la garantie d'un accès facilité à ce genre de soins essentiels dans la vie d'une femme, qu'il s'agisse de régler des questions purement sanitaires, des questions de sexualité ou de maternité.

la prise en charge des examens de gynécologie médicale pour les mineures. Cette mesure pourrait être financée par la création d'une contribution additionnelle pour les entreprises assurant l'exploitation en France

alors que celui-ci bénéficie aujourd'hui à toutes les assurées mineures, quel que soit leur âge. Cette restriction d'âge ne me paraît pas opportune. De plus, je rappelle que le tiers payant est déjà largement pratiqué dans les établissements de santé. En outre, le financement de cet amendement repose sur la création d'une taxe additionnelle à la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques,

afin de les encourager à s'installer dans les zones sous-denses. En effet, l'augmentation du nombre de déserts médicaux témoigne de l'inefficacité des politiques qui ont été mises en oeuvre jusqu'à présent. Un nombre préoccupant de Français rencontrent des difficultés à accéder aux soins dans des conditions de proximité et de délais satisfaisantes. Nous devons aujourd'hui instaurer des règles de régulation territoriale pour l'installation des médecins, à l'instar de ce qui existe déjà pour de nombreuses autres professions de santé, car, si la télémédecine présente des avantages, elle ne saurait faire office de palliatif lorsque le manque de praticiens se fait criant dans les territoires. un dispositif prévoyant que dans les zones dans lesquelles existe un fort excédent en matière d'offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s'installer en étant conventionné à l'assurance maladie que lorsqu'un médecin libéral de la même zone cesse son activité. son activité. Ce dispositif ne s'appliquerait pas aux médecins qui souhaitent conventionner avec l'assurance maladie en secteur 1 dans un territoire où l'offre de soins est abondante et où les médecins conventionnés en secteur 2 sont nombreux. Nous préconisons donc, au travers de cet amendement, une réforme claire de l'installation des médecins libéraux par la mise en place de règles de régulation territoriale efficaces.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Une note récente de Bercy souligne que le nombre de médecins qui choisissent la voie libérale n'est pas compensé par le nombre d'étudiants formés depuis la suppression, en mars dernier,

malgré les différentes mesures incitatives d'installation, comme les aides financières mises en place depuis 2013 pour inciter les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Les différentes incitations n'ont pas eu d'effet sur ces déserts médicaux. Si une adaptation temporaire et ciblée du principe de libre installation dans les zones particulièrement surdotées

de médecins, pour leurs forts excédents en matière d'offre de soins, un nouveau médecin libéral ne puisse s'installer en étant conventionné que lorsqu'un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le conventionnement ne serait plus possible

Certains des dispositifs proposés passent par la voie conventionnelle pour instaurer ce conventionnement sélectif ; d'autres passent par les agences régionales de santé, directement ou à défaut d'accord conventionnel. Le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales, s'était déjà opposé, lors de la discussion de la loi Santé en 2019, aux mesures de restriction à la libre installation des médecins libéraux sur le territoire, car ces mesures sont de faible efficacité.

qu'ils fonctionnent. Les jeunes médecins sont attachés à l'attractivité d'un territoire et aux conditions d'exercice, notamment à l'exercice regroupé. Ils sont de plus en plus demandeurs du salariat,

vote. Tout comme vous, je trouve inacceptable que certains Français soient éloignés de l'accès à la santé. Néanmoins, je crois que les solutions que vous proposez ne sont pas les bonnes. J'ai eu l'occasion de m'intéresser à ce sujet,

Je trouve scandaleux que vous puissiez reprocher à un étudiant en médecine de coûter à l'État 150 000 euros.

des professionnels de santé libéraux, qui ont été évoquées. Il s'agit de faire en sorte que ces professionnels de santé puissent avoir, dans les règles conventionnelles, de quoi prendre en charge le congé de paternité, de maternité ou le congé d'adoption. L'avenant n° 3 de la convention médicale a instauré une aide financière complémentaire à destination des médecins libéraux interrompant leur activité pour cause de maternité, de paternité ou de congé d'adoption, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion du cabinet médical. Mais l'arrêt d'activité rend difficile la prise en charge d'un cabinet. Actuellement, les praticiennes libérales paramédicales perçoivent une indemnité journalière de 56,35 euros, ainsi qu'une allocation forfaitaire unique de repos maternel de 3 428 euros

de la commission ? Ces amendements ont pour objet la possibilité, dans le cadre des négociations conventionnelles, d'accorder une aide financière supplémentaire aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux se trouvant en congé pour cause de maternité ou de paternité. Cet avantage a été accordé aux médecins libéraux en 2017, par la voie d'un avenant à la convention médicale. Les médecins bénéficient ainsi d'une aide financière pour maternité, paternité ou adoption, en complément des indemnités journalières auxquelles ils sont éligibles. Il me paraît donc souhaitable d'ouvrir cette possibilité pour ces professionnels de santé dans le cadre des négociations conventionnelles. La commission émet donc un avis favorable sur ces deux amendements sénateurs, vous demandez l'extension de l'aide complémentaire maternité aux auxiliaires médicaux et aux sages-femmes conventionnées. Je rappelle toutefois que des aides financières existent déjà pour les congés maternité ou paternité de ces professionnels. Les professionnels de santé libéraux peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire de 3 377 euros et d'indemnités journalières forfaitaires.

16 semaines pour une naissance simple. Ces dispositifs permettent d'obtenir des taux de remplacement de leurs revenus importants, compris, en moyenne, entre 82 % et 145 % en fonction des professions paramédicales et sages-femmes.